... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je renouvelle à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs voeux pour cette année

Qu'elles soient légitimes et généreuses, souvent contradictoires ou irréalistes et parfois provocatrices, les revendications exprimées doivent être écoutées. Toutefois, elles ne sauraient en aucun cas justifier le déferlement de violences, de menaces, d'invectives et de dégradations que subit notre pays depuis mi-novembre. Le bilan humain dramatique- 10 morts et plus de 2 500 blessés -devrait un peu plus interroger les acteurs de ce mouvement et ceux qui l'ont soutenu avec parfois un objectif malsain de récupération. Je tiens ici, au nom du groupe du RDSE, à renouveler tous nos remerciements et notre soutien aux forces de l'ordre, aux personnels de santé et aux services d'urgence, très sollicités pendant cette période. Sur le plan économique et social, cet épisode a flétri l'image, et donc l'attractivité, de notre pays et a été destructeur d'activités et d'emplois. Au-delà des mesures très significatives- 10 milliards d'euros -que vous avez annoncées et qui ont été votées courant décembre par l'Assemblée nationale et le Sénat, le débat national, engagé avant-hier, va s'enrichir de propositions concernant, en particulier, la démocratie de proximité, les services publics, la fiscalité et le pouvoir d'achat. Ce grand débat va susciter beaucoup d'espoirs, qu'il ne faudra pas décevoir. À côté de réformes structurelles plus longues à mettre en place, des mesures concrètes d'application immédiate seront attendues par nos concitoyens. Comment envisagez-vous d'y répondre, dans quels domaines et selon quel calendrier ? ? Pensez-vous associer le Parlement, en particulier le Sénat, représentant des territoires, à l'élaboration de ces mesures et de ces réformes, en amont d'un examen strictement législatif des projets de loi ? La parole

Mutilés, éborgnés, défigurés, subissant quotidiennement la violence symbolique et sociale imposée par les politiques gouvernementales, c'est désormais dans leur chair que sont frappés de nombreux « gilets jaunes Face à cette crise majeure et à des rassemblements protestataires, qui ne sont certes pas exempts, parfois, de violences, l'unique réponse apportée par l'exécutif est une répression disproportionnée plus de 5 600 interpellations et gardes à vue, plus de 1 000 condamnations ; on recense 3 000 blessés, dont 94 graves. Les violences policières vont avec l'usage d'armes toujours plus dangereuses : grenades de désencerclement, flash-ball et autres LBD 40, sans oublier le tabassage et le gazage quasi systématique.

Ma question est simple : n'est-il pas temps de mettre un terme à cette répression d'une brutalité intolérable et d'interdire, comme le préconise le Défenseur des droits, l'utilisation d'armes non létales par les forces de l'ordre

nous allons entrer dans le grand débat lancé par le Président de la République. Comme nous l'avons déjà dit publiquement, les parlementaires socialistes en prendront toute leur part sur le terrain, dans les communes. Nous sommes de fervents défenseurs du dialogue et du débat politique avec les Français. Nous répéterons, à cette occasion, les propositions que nous avons déjà faites et que vous n'avez malheureusement pas suivies. Il en est une, toutefois, dont nous ne savons plus si nous aurons le droit de la formuler. Je veux parler, bien sûr, du rétablissement de l'ISF. Le Président de la République a soufflé le chaud et le froid sur ce point. Qui devons-nous croire ? Le Président de, qui exclut toute remise en cause de sa ligne économique et sociale, ou celui du débat en Normandie, qui ouvre le droit à parler de l'ISF ? Ce sujet pose plus largement la question de la prise en compte de la parole des Français dans ce débat, à l'image de vos reculs contraints sur une partie de l'augmentation de la CSG pour les retraités, sur la taxe carbone, sur le coup de pouce au SMIC la prime d'activité et, désormais, sur vos 80 kilomètres par heure. Entendez-vous infléchir votre politique économique et sociale si contestée ou ce débat ne sera-t-il qu'un exercice de communication sans suite ? Enfin, monsieur le Premier ministre, permettez-moi une dernière question : comment envisagez-vous la conclusion de ce grand débat ? Accepterez-vous, comme vous l'ont demandé certains syndicats, qu'elle prenne la forme d'une vraie négociation avec les partenaires sociaux, que vous avez négligés jusqu'ici ?

mais pour dire quel est le cadre dans lequel nous allons prendre en compte ce que diront les Français. Je vais vous donner un exemple, qui, parce qu'il est évident, illustrera cette logique. Imaginez- j'espère que ce ne sera pas le cas, évidemment -que les Français veuillent remettre en cause la forme républicaine de nos institutions. Je ne crois pas qu'ils le feront, même si nous devons faire attention à préserver ce qui nous semble parfois acquis.

En répondant à ces questions, en s'exprimant sur ces sujets, les Français vont nous donner un certain nombre d'indications. Il appartiendra ensuite au Gouvernement, au Parlement, à l'ensemble de ceux qui concourent au débat public, d'en faire leur miel, de s'en inspirer, dans la réponse qu'ils apporteront aux questions profondes et anciennes qui taraudent notre société. C'est dans cet esprit que nous nous engageons.

une grande conférence territoriale et sociale qui permettrait à l'ensemble des acteurs d'échanger sur ce qui ressort du grand débat

Si ce débat prospère, comme nous le souhaitons et comme, à mon sens, un très grand nombre de Français l'espère, alors peut-être faudra-t-il faire droit à cette proposition. Je crois qu'il est un peu tôt pour répondre à cette question, car il faut laisser au débat le temps en garantissant aux Français, ainsi que nous l'avons fait, que le Président de la République l'a dit et que je le redis ici, devant les sénateurs, que nous tiendrons compte des éléments qui seront formulés à l'intérieur du cadre proposé par le Président de la République. Monsieur le Premier ministre, j'entends votre réponse et je vous confirme que les parlementaires socialistes participeront au grand débat national qui a été lancé par le Président de la République. La démocratie participative peut enrichir la démocratie représentative,

Le 15 décembre dernier, un navire de pêche était intercepté au large de La Réunion avec, à son bord, près de soixante-dix personnes, dont des femmes et des enfants, originaires du Sri Lanka.

Ces faits laissent penser qu'une nouvelle filière est en train de se structurer pour fuir la crise politique, ethnique et religieuse qui divise l'ancien Ceylan. Dix ans après la fin de la guerre civile, qui causa la mort de près de 100 000 personnes, les minorités tamoule et chrétienne restent en proie aux persécutions. La Réunion représente une porte d'entrée vers la France, pays des droits de l'homme, où la diaspora sri-lankaise est évaluée à environ 150 000 personnes. Sur les quelque quatre-vingts migrants qui ont rejoint notre île en l'espace de dix mois, certains ont formulé des demandes d'asile, d'autres ont déjà été reconduits chez eux, avec les conséquences que l'on peut imaginer. En plus de nous alerter sur le drame humain que vit cette population, l'ouverture de cette nouvelle voie migratoire vers La Réunion suscite de vives inquiétudes dans la population. population. Monsieur le ministre, les autorités disposent-elles de moyens adéquats pour assurer la surveillance des côtes réunionnaises ? Quelle position le Gouvernement compte-t-il adopter face à ce phénomène aussi soudain qu'inattendu qui touche La Réunion ?

Monsieur le sénateur, je vous confirme que, depuis le mois de mars de l'année dernière, nous avons enregistré l'arrivée de quatre navires sur les côtes réunionnaises, transportant un certain nombre de personnes qui auront donc fait un périple de plus de 4 000 kilomètres

d'éviter que ne se reconstitue une filière d'immigration clandestine du Sri Lanka vers La Réunion, qui serait, au final, une nouvelle filière de traite des êtres humains. La Monsieur le Premier ministre, dans le livre, qu'il a publié juste avant d'être élu Président de la République, Emmanuel Macron écrivait : « Aujourd'hui, les Français ont l'impression que leurs gouvernements ne gouvernent plus. L'Europe, les partis, les marchés, les sondages, la rue, il existe une confusion sur le détenteur du pouvoir. Quand il n'y a pas de clarté du Gouvernement, le peuple se cabre. Il faut savoir expliquer plutôt que de faire de la communication. Une nouvelle étape de la déconcentration de l'État est nécessaire. Je crois dans un nouveau partage démocratique. C'est le fondement de la République contractuelle dont nous avons besoin, la République qui fait confiance aux territoires, à la société et aux acteurs pour se transformer. Les collectivités locales et leurs élus doivent jouer un rôle accru. C'est une nouvelle étape de transfert des pouvoirs vers ces collectivités que nous devons décider. » Excellent texte ! Nous ne saurions mieux dire, monsieur le Premier ministre la crise des « gilets jaunes » se traduit par une rupture brutale du lien de confiance entre le peuple, le Président et son gouvernement, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, depuis deux ans, le Président de la République fait très exactement le contraire de ce que préconisait le candidat Macron, en recentralisant à outrance et toujours plus, en rejetant le rôle prééminent des maires, que vous prenez subitement en considération ? Êtes-vous enfin prêt à mettre en oeuvre les conditions d'une déconcentration de l'État, comme vous le disiez, ainsi qu'une nouvelle étape de décentralisation massive et d'expérimentation en faisant confiance aux élus locaux et aux partenaires sociaux, comme vous le demande, dans les conférences, le président du Sénat, garant, aux termes de la Constitution, de l'équilibre des pouvoirs et des territoires ? Bref, êtes-vous prêt à changer radicalement de méthode en agissant du bas vers le haut et non plus du haut vers le bas, pour éviter que votre grand débat ne se transforme en grande débâcle ?

Monsieur le ministre, vous l'aurez compris au vu de ce que j'ai lu, nous préférons les preuves d'amour aux déclarations d'amour. Nous attendons une grande conférence territoriale et une grande conférence sociale après le grand débat. Nous attendons une loi de décentralisation et nous attendons que vous mettiez en pratique les choses en respectant le Sénat,

Les Français regardent les sociétés d'autoroutes avec suspicion, et pour cause ! Si la qualité de service y est globalement élevée, les tarifs le sont aussi, ce qui est inversement proportionnel à la transparence financière qui régit cet oligopole. Depuis les conditions de privatisation très discutables de 2005, ces sociétés prétendent ne pas gagner beaucoup d'argent. Elles nous en feraient presque pleurer ! Pourtant, elles ne savent pas quoi inventer pour demander aux gouvernements successifs d'allonger les durées des concessions. Malheureusement, l'État désargenté cède à chaque fois aux mirages de travaux plus ou moins utiles- réalisés par les propres filiales contre quelques années encore de punition tarifaire pour les automobilistes. Et ne parlons même pas des turpitudes électoralistes d'une ministre du précédent quinquennat qui vont conduire à alourdir de nouveau la facture dès le 1 février À l'heure où les Français veulent retrouver du pouvoir d'achat et exigent plus de transparence, il est temps de faire la lumière sur cette situation. Ces sociétés seraient prêtes, prétendument, à faire un geste, mais nous n'en connaissons pas les conditions financières et nous ne sommes donc pas capables d'apprécier si l'effort envisagé est réel ou s'il s'agit d'une aumône presque insultante. Le Gouvernement étudie actuellement ces propositions. À partir de quel niveau les jugera-t-il acceptables ? Les sociétés d'autoroutes abandonneront-elles 20 %, 30 % ou 50 % des augmentations prévues ? Il semble aussi que leur lobbying soit intense pour prendre en charge de nouvelles sections d'autoroute, contre un allégement de la durée des concessions. Qu'en est-il ? Pouvez-vous nous assurer que les discussions seront menées sans opacité et en prenant en compte la réelle situation financière de ces sociétés ?

19 kilos de cocaïne ont été retrouvés dans les bagages d'une mère et de ses enfants à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne. Voilà le quotidien des Guyanais En quelques années seulement, la Guyane, terre d'Amérique du Sud, est devenue un espace majeur de transit vers l'Europe. Imaginez que, entre 2014 et 2018, les saisies ont augmenté de 335 passant de 145 à 631 kilogrammes ! Si bien que, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, près de 30 % du marché français, évalué entre 25 et 30 tonnes, proviendrait de la Guyane. Concrètement, on compterait de 20 à 30 « mules » par avion, soit plus de 3 000 personnes par an, dont seulement 10 % sont interpellées. À l'origine de ce trafic, un ennemi sans visage, qui se cache derrière le destin tragique de ces « mules », qui transportent la drogue dans leurs bagages, quand elles ne l'ingurgitent pas au péril de leur vie.

Parce que la société n'est aujourd'hui pas en mesure de leur proposer un emploi, de leur offrir un avenir, ces jeunes risquent volontiers leur vie contre le mirage de quelques milliers d'euros.

que le trafic s'accroît considérablement et, avec lui, le nombre de ses victimes. C'est pourquoi je vous le demande solennellement : le Gouvernement entend-il déployer un plan ambitieux de prévention et de lutte contre le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane ? La parole

Le 30 décembre dernier, pour les fêtes de fin d'année, est paru un décret d'application de la loi joliment intitulée « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », un décret visant à renforcer le contrôle des chômeurs, dans l'idée que les Français les plus fragiles seraient responsables de leur exclusion. Voici donc comment ce décret entend responsabiliser « ceux qui déconnent », qui « n'ont pas le sens de l'effort », selon les termes choquants employés sans vergogne par le Président de la République : dès le premier refus d'une offre, le chercheur d'emploi pourra être radié des listes de Pôle emploi ; l'offre raisonnable d'emploi est redéfinie, le salaire précédent n'étant plus un motif de refus

les syndicats ont fortement réagi contre ce nouveau caporalisme déshumanisé visant les demandeurs d'emploi. On ne peut pas vouloir baisser le chômage en radiant les allocataires ou en accroissant la précarité des exclus de l'emploi. En raison de la masse des dossiers suivis et de l'explosion des CDD de moins d'un mois, les agents de Pôle emploi estiment que ce climat de suspicion dénature leur mission. Sans compter que vous avez supprimé 800 postes dans la dernière loi de finances Ne serait-il pas temps, madame la ministre, à l'heure où vous semblez vouloir adopter une autre attitude à l'égard des syndicats et en vue du grand débat, de modifier votre analyse de la situation de l'emploi, de privilégier enfin l'accompagnement des précaires de questionner non seulement l'employabilité des personnes, mais aussi le nombre et la qualité des emplois proposés par les entreprises

madame la ministre, vous poursuivez une logique technocratique et ajoutez de la culpabilité à la précarité. Vous mettez en danger une population déjà affectée par le sentiment d'injustice. Vous n'avez pas écouté la réponse ! Ce décret est de très mauvais augure en vue de la réforme systémique de l'assurance chômage actuellement sur la table des négociations.

Vous connaissez ma conviction sur le sujet : j'estime que cet impôt doit être supprimé pour l'ensemble des ménages. Cela n'exclut pas que la question soit posée aux Français, mais je vous rappelle ma position. Très bien ! S'agissant de l'impôt sur la fortune et du prélèvement forfaitaire unique, je réaffirme cette conviction forte : il faut baisser l'impôt sur le capital pour que nos entreprises puissent investir, innover et créer des emplois.

vingt ans que l'on fait croire aux Français qu'on peut avoir une industrie forte avec des impôts élevés. Le million d'emplois supprimés dans l'industrie montre que ce n'est pas la bonne voie. Nous poursuivrons donc la baisse des impôts sur l'industrie

ans n'empêche pas d'aller chercher l'argent là où il se trouve en mettant en place, comme nous allons le faire, une juste taxe sur les géants du numérique, qui s'appliquera à compter du 1 janvier 2019, pour que tous les géants du numérique payent en France le même montant d'impôt que nos PME ! Très bien ! La parole

écologique et solidaire, j'appelle votre attention sur la création et l'exploitation d'une retenue d'eau collective, le lac de Caussade, en Lot-et-Garonne. Il s'agit d'un lac collinaire de moins de un million de mètres cubes, destiné à l'irrigation. La réalisation de ce lac serait pour les agriculteurs un espoir : une partie des eaux de pluie hivernales pourrait être stockée pour être utilisée en période estivale. Ce serait aussi une opportunité de maintenir un étiage convenable du petit ruisseau en aval de la retenue pendant l'été. Les porteurs de projets dans le monde agricole, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs, se heurtent à des textes qui rendent quasiment impossible la réalisation de telles opérations. C'est peut-être cette complexité des lois et des normes qui a poussé les agriculteurs à enfreindre la loi et à entreprendre la construction de l'ouvrage, solution que je déplore mais qui est une réalité.

Je vous demande donc quelles mesures vous envisagez de prendre pour résoudre ce problème et permettre une sortie par le haut. Vous le savez comme moi, le changement climatique est malheureusement en marche, et le monde rural va connaître des sécheresses de plus en plus graves. Aussi, envisagez-vous d'adapter la loi sur l'eau afin de mieux répondre aux défis majeurs qui nous attendent ?

la question du stockage de l'eau- il faut bien appeler les choses par leur nom. S'agissant de la situation à Caussade, je tiens à rappeler que les défenseurs pu apporter la preuve de sa compatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le fameux SAGE que tous les élus locaux connaissent bien, et avec les directives européennes en vigueur,

contre l'avis de deux préfets de région. Nous en avons d'ailleurs tiré les conséquences en ce qui concerne la préfecture de département. Malgré ce retrait, le projet a été lancé illégalement

La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. » Ainsi parlait Victor Hugo, l'un de nos éminents devanciers. cet édifice commun est aujourd'hui trop souvent attaqué. Inadmissibles, les agressions répétées de journalistes mettent en danger le pacte républicain ! En s'attaquant à la presse, en bloquant la diffusion de journaux, en menaçant une journaliste de viol, comme à Toulouse, des insultes sur les réseaux sociaux, c'est la République que l'on agresse. Mais personne ne tordra le bras à la République. La France n'acceptera jamais de banaliser le bâillon Ailleurs, la liberté de la presse est peut-être un luxe ou une chimère. En France, c'est un droit fondamental d'informer, de créer le débat, de divertir. N'oublions pas que, dans le monde,

la meilleure façon d'honorer nos morts est de défendre, sur le terrain comme en ligne, la liberté de la presse et le travail des journalistes.

Sans cette liberté, sans les médias, sans les journalistes et leur travail, il n'y a pas démocratie possible. Les journalistes sont les vigies de la démocratie, et une démocratie qui ne défend pas sa presse est une démocratie qui s'oublie, une démocratie qui se nuit Le journaliste peut évidemment être contesté, critiqué ; il doit bien sûr faire l'objet de controverses et il doit aussi rendre des comptes. Mais rien ne justifie les appels à la défiance, puis à la haine, puis à la violence, que nous avons entendus. Rien ne justifiera que l'on cherche, par la force ou par la peur, à bâillonner les uns ou les autres. Dans ce débat qui nous occupe, où les journalistes sont de plus en plus souvent mis en cause, il est une arme essentielle : l'éducation aux médias. Nous ne ménageons pas nos efforts en Le traitement de l'information appelle aussi l'exigence déontologique la plus forte. C'est pourquoi le Gouvernement a confié une mission à Emmanuel Hoog, qui procède depuis quelques semaines à la concertation la plus large possible sur le sujet, pour aboutir à des propositions. Défendre la liberté de la presse, c'est aussi lutter contre les tentatives de manipulation de l'information

deux assemblées. Défendre la liberté de la presse, c'est rendre possible la diffusion des idées sur tout le territoire. C'est pour cela que nous prenons à bras-le-corps la question de la distribution de la presse

Je crois au bicamérisme, qui garantit une démocratie mieux équilibrée. Il n'est pas de République forte sans institutions puissantes. Nées de temps troublés, nos institutions sont résistantes aux crises et aux turbulences. » Sans doute, monsieur le Premier ministre, aurez-vous reconnu les mots d'Emmanuel Macron, Président de la République, le Congrès en juillet 2017 et en juillet 2018. Il avait raison : nous connaissons une crise sociale, une crise culturelle, une crise territoriale, mais nous ne connaissons pas de crise des institutions. Eh oui ! Pourtant, dans sa, le Président de la République met en discussion la transformation du Sénat. quelles sont vos intentions à l'égard de notre

du dialogue permanent entre deux assemblées tirant leur légitimité de modes de désignation et de temporalités différents. C'est un élément constitutif de notre de notre équilibre démocratique. Il n'est d'ailleurs pas propre au génie français, même si celui-ci est considérable, puisque, dans toutes les démocraties, c'est ce dialogue

Le Président de la République, dans le débat qu'il a engagé, a ouvert un chapitre sur la démocratie et la citoyenneté.

à faire en sorte que nos institutions fonctionnent mieux, que notre bicamérisme fonctionne mieux et que nos concitoyens soient toujours convaincus qu'il fonctionne comme il devrait fonctionner. Tel est le sens du débat : je crois que ces questions sont très raisonnables et intéressent nos concitoyens.

Lorsqu'il veut prendre des mesures contre les casseurs, il reprend la proposition de loi du président Retailleau. Avant de songer à transformer le Sénat, peut-être l'exécutif devrait-il songer à transformer son regard sur le Sénat. Nous ne sommes pas qu'un contre-pouvoir encombrant ; nous sommes aussi et avant tout la voix des territoires de France

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, chaque samedi depuis maintenant deux mois, en marge des manifestations des « gilets jaunes », un certain nombre de centres-villes de notre pays sont le théâtre de violences et d'affrontements inacceptables. On ne compte plus les commerçants, artisans, membres des professions libérales qui ont vu leurs locaux attaqués, dégradés ou pillés. Quant à ceux qui ont eu la chance d'échapper à ce déchaînement gratuit de haine, ils vivent dans l'angoisse des samedis à venir et constatent de semaine en semaine, la mort dans l'âme, le déclin de leur activité. Craignant pour leur sécurité, les clients délaissent en effet massivement les centres-villes. Chiffre d'affaires en baisse de plus de 40 %, chômage technique, licenciements constituent aujourd'hui le lot quotidien de nos commerçants, artisans, restaurateurs et hôteliers. hôteliers. Si rien ne change, si rien n'est fait pour les soutenir, on assistera très probablement à une explosion du nombre des dépôts de bilan. Or, monsieur le ministre, ces commerçants et ces artisans jouent un rôle non seulement économique, mais aussi social. Plusieurs municipalités, conscientes qu'il ne peut y avoir de centre-ville sans commerces, vont prendre des mesures d'urgence. C'est le cas de Toulouse, où un conseil municipal exceptionnel examinera un plan d'aide de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais les communes ne peuvent pas tout : les maires prennent leurs responsabilités ; l'État doit également prendre les siennes ! Plusieurs propositions d'aides individualisées seront formulées, notamment l'exonération, et non le simple report, des charges sociales patronales pour les mois de décembre l'exonération de la CFE, ainsi que le report de la mise en application de la révision des valeurs locatives commerciales. Monsieur le ministre, entendez-vous le désespoir des commerçants et artisans des centres-villes ? Comptez-vous leur venir en aide ? C'est urgent

qui ont été le plus touchés. Nous restons en permanence ouverts au dialogue avec les représentants des commerçants et des artisans. Je vous confirme également que nous avons demandé aux assureurs de répondre le plus rapidement possible aux difficultés des commerçants.

européenne. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Or, aujourd'hui, plus de deux ans et demi après le référendum du 23 juin 2016 et à soixante-dix jours à peine de l'échéance du 29 mars, force est de constater que rares sont ceux à qui cette évidence apparaît encore et qui savent ce que le Brexit signifiera réellement. La seule certitude qui se dessine chaque jour plus clairement est que le Brexit sera tout sauf la marche glorieuse vers la liberté et l'Eldorado que certains avaient promis. Quelle que soit la forme qu'il prendra, il ne fera en définitive que des perdants, au Royaume-Uni comme dans le reste de l'Europe. Le brouillard qui entoure le processus de retrait demeure et s'est même encore épaissi. Il avait pourtant semblé un peu se dissiper en novembre dernier avec la conclusion, après dix-sept mois de laborieuses négociations, d'un accord de retrait et une déclaration politique esquissant les grandes lignes des futures relations entre le Royaume-Uni et le continent. Je tiens à cet égard à saluer une nouvelle fois l'action de mon collègue des pays de Savoie Michel Barnier, qui a su admirablement maintenir l'unité des Vingt-Sept tout au long des discussions, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Le texte qu'il a négocié était peut-être imparfait ; comment aurait-il pu d'ailleurs en être autrement avec un gouvernement britannique prisonnier de ses propres contradictions, longtemps incapable d'assumer le fait qu'il lui faudrait bien trancher un jour entre, d'un côté, les exigences des, et, et, de l'autre, la préservation des intérêts économiques du Royaume-Uni et l'absence d'une frontière physique en Irlande ? Si certains ont pu juger la position européenne trop inflexible, insuffisamment pragmatique, il n'en reste pas moins que ce projet d'accord était sans doute le meilleur possible au regard de la complexité de la situation et, bien sûr, de la nécessité de protéger les intérêts de l'Union européenne, au premier chef l'intégrité de son marché unique. Cependant, comme on pouvait malheureusement s'y attendre, en particulier depuis le 10 décembre et le report du, qui n'aura finalement pas eu l'effet escompté, les contradictions britanniques ont resurgi à la Chambre des communes.

Plus que jamais, le processus semble échapper à tous, dans un climat politique de plus en plus dégradé. À ce stade, tous les scénarios restent en théorie ouverts, sauf peut-être celui d'élections générales anticipées, Theresa May ayant, en dépit de son échec cuisant, conservé hier soir la confiance de sa majorité. Mais ses marges de manoeuvre sont désormais extrêmement réduites, d'autant que les Européens ont à plusieurs reprises, et encore hier par la voix de la Commission européenne, exclu toute renégociation du texte finalisé en novembre. Madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer si cette position vous paraît en réalité toujours aussi ferme ? Au regard de la situation actuelle et malgré la lassitude qu'inspire ce feuilleton sans fin, certains États membres pourraient-ils être tentés d'accéder à une demande de renégociation de l'accord de retrait ?

Quant à l'option de la tenue d'un second référendum, bien que fermement écartée par Theresa May, et malgré les désaccords profonds sur la ou les questions à poser dans le cadre de cette nouvelle consultation, elle a repris une vigueur certaine et ne peut plus être exclue. D'autres issues, que nous n'anticipons peut-être pas encore, pourraient également se faire jour. Dans un certain nombre de cas, un report de l'échéance du 29 mars serait vraisemblablement nécessaire. Si un tel cas de figure est bel et bien prévu par l'article 50 du traité de l'Union européenne, comment le concilier avec la tenue au mois de mai prochain des élections européennes, prévues sans représentation du Royaume-Uni et qui ne sauraient être prises en otage par les vicissitudes de la vie politique britannique ? ? Il reste un dernier scénario que je n'ai pas encore évoqué, et qui est peut-être celui qui a le plus pris corps avec le rejet de l'accord de retrait, bien qu'une majorité de députés britanniques affirment s'y opposer. Il s'agit évidemment du scénario du, dont le risque, selon les mots de Michel Barnier, « n'a jamais paru aussi élevé » qu'aujourd'hui. Je note d'ailleurs que le Premier ministre a déclenché le plan destiné à faire face à un Brexit sans accord. d'un est redoutée depuis des mois, l'impression qui domine est que personne jusqu'à maintenant n'a semblé vouloir véritablement y croire. À cet égard, l'état de préparation, ou plutôt de non-préparation, de nos entreprises est significatif. Je ne suis pas non plus convaincu que chacun, en Europe comme au Royaume-Uni, ait tout à fait pris conscience de l'ampleur des implications d'une sortie sans accord, qu'un membre de l'équipe européenne de négociation a récemment qualifiées de « tectoniques

de paiement de sa contribution par le Royaume-Uni, il faudrait trouver pas moins de 10 milliards d'euros en 2019 pour compenser les sommes non versées par Londres entre mars et décembre, et 12 milliards d'euros de plus pour l'ensemble de l'année 2020.

Dans l'hypothèse d'une sortie « sèche » du Royaume-Uni, où aucune période de transition ne trouverait à s'appliquer, c'est presque du jour au lendemain que quarante-cinq ans d'acquis communautaires seraient effacés. Plus aucun lien juridique, plus aucun cadre de coopération autres que ceux qui sont prévus par les accords bilatéraux et multilatéraux ne lieraient dès lors le Royaume-Uni à l'Europe. Le choc d'une telle rupture serait évidemment brutal et ses conséquences seraient aussi innombrables qu'immédiates, même si des mesures de contingence sont en cours de finalisation au Royaume-Uni, au niveau européen et, comme nous le verrons tout à l'heure, au niveau national. Madame la ministre, pourriez-vous nous informer de l'état d'avancement des mesures de préparation proposées par la Commission européenne, mais aussi des éventuels engagements pris par le Royaume-Uni au sujet des droits des citoyens européens en cas de ? Ne de ? Ne nous y trompons cependant pas, ces dispositions ne régleront pas tout et ne remplaceront pas un accord permettant un Brexit aussi ordonné que possible et la construction d'un nouveau partenariat. Elles n'en ont d'ailleurs pas l'ambition. Ce sont ainsi quasiment tous les aspects de notre relation économique et commerciale avec le Royaume-Uni qui, à plus ou moins brève échéance, seraient affectés. Les perturbations qui en résulteraient feraient peser des risques supplémentaires sur la croissance et l'emploi, notamment dans nos territoires qui bordent la Manche, qui se retrouveraient dès lors en première ligne. C'est également tout un pan de notre partenariat en matière sécuritaire et stratégique qui serait mis à bas, alors même que les risques et les menaces planant sur notre continent se font aujourd'hui de plus en plus pressants. Dans un contexte où, après trois ans de débats et de négociations, tant de liens qui nous unissent encore seraient si brusquement rompus, où les échanges humains que nous entretenons se trouveraient nécessairement réduits, je m'interroge sur la capacité des Européens et des Britanniques à retisser rapidement les fils d'une relation solide et de long terme. Pourtant, celle-ci sera demain toujours aussi essentielle pour faire face ensemble aux défis du XXI siècle. La parole

C'est une mauvaise nouvelle, que nous regrettons, d'abord parce que l'accord de retrait que Theresa May a soumis à ratification a été négocié pendant près de deux ans.

Vous le savez, cet accord de retrait et la déclaration politique sur les relations futures avaient fait l'objet d'un accord entre les négociateurs, avant d'être approuvés par les chefs d'État et de Gouvernement des vingt-sept États membres, réunis à l'occasion d'un sommet extraordinaire le 25 novembre dernier.

L'objectif principal était de réduire les incertitudes et de limiter les perturbations provoquées par le retrait, en particulier pour les citoyens, les acteurs économiques et l'ensemble des parties prenantes. Les inquiétudes des parlementaires britanniques conservateurs, notamment, portaient principalement sur le mécanisme de, de « filet de sécurité » pour éviter le rétablissement d'une frontière dure entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord si la nature des relations futures ne l'empêchait pas. Pour y répondre, les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne avaient, en amont du vote, confirmé à Mme May que, conformément aux conclusions du Conseil européen du 13 décembre et aux propos tenus à cette occasion par le Président de la République, le filet de sécurité, s'il devait être activé,

Cela n'aura de toute évidence pas suffi, et le rejet de l'accord, même s'il tient à des raisons différentes selon les bancs, est plus profond. Mme May ayant remporté le vote sur la motion de censure qui a été organisé hier soir à la Chambre des communes, il lui revient de décider des conséquences qu'elle tire de ce rejet et de préciser ses intentions pour les prochaines étapes. Elle le fera dès lundi 21 janvier devant la Chambre des communes, après d'intenses consultations parlementaires dans le cadre d'un processus transpartisan. Si elle parvient à des avancées sur le fond, elle reprendra contact avec la partie européenne. Ce n'est évidemment pas à nous Français, Européens, de dire aux Britanniques ce qu'ils doivent faire.

permettant que le Royaume-Uni, à l'avenir, reste proche de l'Union européenne, est connu : c'est la ratification de l'accord de retrait. La plus grande incertitude pèse aujourd'hui sur les intentions britanniques. Aucune option ne peut être théoriquement exclue, y compris une demande de report de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Celui-ci est juridiquement et techniquement possible,

quelle échéance ? En vue de quel type d'accord ? Avec quelles garanties que cette demande recueillera le soutien d'une majorité des parlementaires britanniques ? À quoi servirait, sinon, un report de quelques semaines ou de quelques mois, qui poserait la question délicate et baroque du mode de désignation de députés européens britanniques au parlement de Strasbourg ? Un report aurait cependant du sens par exemple pour finaliser la ratification d'un accord de retrait, ou encore si le Royaume-Uni évoquait la possibilité de rester dans l'Union européenne. Notre porte reste bien entendu grande ouverte, mais la vérité oblige à dire qu'à ce stade scénario de politique-fiction, que rien ne vient conforter de la part du Gouvernement britannique. Dans ce contexte délicat, deux points me semblent importants.

resterait néanmoins préférable à un mauvais accord, qui ne respecterait pas l'intégrité du marché unique ou ne fournirait pas le « filet de sécurité » dont un pays comme l'Irlande a besoin. Le second point, c'est donc que nous devons, plus que jamais, nous préparer à un retrait sans accord, à la fois au niveau européen et au niveau national. Au niveau européen, les travaux préparatoires à une absence d'accord se sont accélérés à partir du mois de novembre 2018. La Commission a publié deux communications sur ce sujet, les 13 novembre et 19 décembre, ainsi que seize propositions de textes législatifs dans différents domaines : visas, efficacité énergétique, services financiers, transport aérien, transport routier, contrôles douaniers, climat, coopération régionale sur l'île d'Irlande, statistiques. Au niveau français, vous le savez, nous avons également accru notre travail de préparation, avec le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnances que je vous ai présenté en novembre. J'espère que ce texte sera tout à l'heure définitivement adopté dans votre hémicycle, ce qui permettra au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que nous soyons prêts, même en l'absence d'accord.

les entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni ou celles qui, installées en France et employant des Français, sont cependant de droit britannique n'aient pas à subir de trop lourdes conséquences d'une absence d'accord.

Nous le savons tous, le programme Erasmus, dont on a fêté récemment le trentième anniversaire, est l'un des grands succès de l'Union européenne, si ce n'est le plus grand, en tout cas le plus visible d'entre eux, d'une portée symbolique forte.

Les étudiants européens seront, quant à eux, privés d'un passage par les établissements britanniques, très réputés. Ils seront traités comme des étudiants internationaux et tenus de payer les frais d'études élevés propres aux établissements britanniques. Heureusement, Erasmus est ouvert à de nombreux pays non membres de l'Union européenne, comme la Norvège, l'Islande ou la Turquie. Il conviendrait donc que les négociations prévoient le maintien de cet avantage précieux pour notre jeunesse. Cela permettrait aussi de restaurer le lien entre les nouvelles générations du Royaume-Uni et de l'Union européenne, lien qui a été rompu sur la base de nombreux mensonges et manipulations politiques. Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que nos étudiants, tout comme ceux du Royaume-Uni, pourront continuer à bénéficier dans des conditions similaires du programme Erasmus ? La parole est à Mme la ministre.

À court terme, nous nous attendons à ce que toutes les mobilités en cours continuent jusqu'à leur terme. Cela implique notamment la poursuite du versement des bourses de mobilité, qui sont attribuées par les universités d'origine des étudiants, donc par les universités françaises, et ne sont pas affectées par le Brexit.

La Commission européenne propose, avec raison, que soit respectée une forme d'équilibre financier entre les contributions et les bénéfices retirés par un État tiers, alors que cette contrainte ne s'applique pas un État membre. Au-delà du programme Erasmus, le Gouvernement britannique s'est engagé à maintenir les frais de scolarité des ressortissants européens au niveau de celui des Britanniques pour l'année 2019-2020, qu'il y ait accord ou non, y compris pour les étudiants qui commenceraient leurs études à la rentrée de 2019. En revanche, il n'a pas pris d'engagement au-delà de 2020.

éventuel retour à des barrières tarifaires. Une partie de notre équipe de direction est française et s'inquiète pour son sort, de même que nombre de travailleurs de notre usine.

notamment parce que nous rencontrons régulièrement, avec Agnès Pannier-Runacher, les fédérations professionnelles et les entreprises. Les préfets en font autant dans les territoires. Je suis d'accord avec vous

La rapidité et la simplicité des démarches administratives sont essentielles pour maintenir l'attractivité de nos départements et, plus largement, pour garantir la viabilité des aéroports de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie.

autorités britanniques. Quelles mesures concrètes le Gouvernement entend-il adopter pour garantir les droits fondamentaux des citoyens britanniques sur notre territoire ? La parole

Nous devons simplifier autant que possible les contrôles qui seront effectués à l'entrée sur notre territoire et nous avons augmenté le nombre d'agents chargés de ces contrôles,

Depuis deux ans déjà, le trafic transmanche du port de Dunkerque connaît une baisse suffisamment sérieuse pour nous inquiéter. La situation risque de s'aggraver encore si les investissements nécessaires à la fluidification du trafic ne sont pas réalisés. Nous pouvons déjà nous féliciter de la construction d'un parking dédié de 200 places et de la construction d'infrastructures pour les contrôles, mais tout semble indiquer que davantage d'investissements

autre sujet d'inquiétude. Les eaux poissonneuses du Royaume-Uni sont les plus étendues d'Europe. Le soutien massif des pêcheurs britanniques au Brexit tenait tant à une contestation des quotas de pêche européens qu'à la concurrence des pêcheurs étrangers, notamment français.

la perspective d'une sortie franche de l'Union européenne- toujours possible -risque de remettre en cause le principe d'un accès peu régulé aux eaux britanniques. Cela nuirait fortement aux pêcheurs français, mais aussi au secteur commercial,

S'agissant des ports, en cas de Brexit sans accord, il sera évidemment nécessaire de rétablir des contrôles, et donc de réaliser les investissements nécessaires pour la construction d'infrastructures. Nous avons recruté

dans quelle mesure les ports français pouvaient être intégrés au corridor mer du Nord-Méditerranée. C'est déjà le cas pour Calais et Dunkerque ; ce le sera pour Le Havre. Le Parlement européen, de son côté, a proposé d'élargir la liste des ports éligibles en

de flécher ce reliquat vers la construction d'infrastructures nécessaires aux ports pour faire face aux conséquences d'un Brexit sans accord. Pour autant, il faut que les gestionnaires des ports candidatent et soumettent

le Royaume-Uni n'ayant pas clarifié sa position pour le moment. Sortir de l'Union européenne ne se fait pas d'un trait de stylo sur un bout de papier ! Toutes les théories fumeuses exploitées par des intervenants politiques en mal de notoriété s'effondrent dès lors que l'on se penche sur les conséquences du Brexit. quitter de l'Union européenne sans dégâts est illusoire. Les effets d'une sortie de l'Union européenne sont redoutables pour l'ensemble de nos concitoyens : elle emporte des conséquences négatives sur le quotidien des expatriés, des entreprises, des travailleurs, des consommateurs. Tout le monde est concerné Le risque d'une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne est aujourd'hui tangible. Même si un report du Brexit est possible, rien ne tend vers un accord durable. Ne règne que le chaos dans lequel les populistes laissent les élus-

mais, désormais, nous devons aussi défendre très concrètement l'Europe face à celles et ceux qui appellent au repli sur soi. Nous savons que les populistes peuvent remporter un référendum, à force de, de coups de menton, d'effets de manche et autres mensonges. Mais, une fois le vote passé et les caméras éteintes, ils ne laissent qu'un amas de problèmes sans solution. Ils ne sont plus là, dès lors qu'il faut agir pour nos concitoyens. Oui, une autre politique pour l'Union européenne, plus juste, plus sociale, plus simple parfois, plus proche des citoyens, L'absence d'Europe n'est pas une alternative crédible. L'absence d'Europe, ce sont des heures d'attente aux postes-frontière, des papiers supplémentaires à remplir pour se déplacer, des diplômes qui ne sont plus reconnus, des entreprises qui ne peuvent plus produire et faire circuler leurs marchandises

est de détruire le projet européen. Souvenons-vous de Nigel Farage, qui proclamait que son premier objectif était de sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, son deuxième de détruire l'Union européenne. Ne l'oublions jamais, et restons déterminés ! Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour faciliter une issue positive du côté britannique ?

le gouvernement de Theresa May et Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, ont posé les bases d'une sortie négociée du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'accord trouvé vient d'être sèchement rejeté par les députés britanniques. Nous constatons que la fracture révélée outre-Manche par le référendum du 23 juin 2016 n'a cessé de se creuser.

Je veux tirer un enseignement de ce triste feuilleton pour tous ceux qui croient aux vertus de la construction européenne. La situation britannique est un révélateur de la fragilité de tout notre édifice européen.

Est-il sérieux d'ouvrir des négociations d'adhésion avec deux nouveaux pays, l'Albanie et la Macédoine, alors que le dossier britannique n'est pas clos et que de nombreuses questions restent en suspens ? Nous devons sauver l'Europe d'elle-même et de ses dérives réglementaires. Nous devons nous montrer à la hauteur des défis de la construction européenne, sans céder aux sirènes du populisme, porteur d'inquiétantes pulsions nationalistes. Soyons responsables et osons rappeler que l'Europe nous apporte plus qu'elle ne nous coûte. Madame la ministre, alors que nous ne pouvons dire avec certitude quels seront les effets concrets du Brexit,

vers l'Union européenne. Cependant, nous le savons, toutes les solutions nécessaires n'ont pas été trouvées, et un certain nombre de médicaments d'importance stratégique, destinés notamment au traitement des cancers de la prostate ou du sein, pourraient ne plus être acceptés par l'Union européenne, ce qui conduirait à une interruption de l'approvisionnement pour plus de 70 000 patients,

en France, que nous souhaitons absolument garder. Que faire pour, de manière pragmatique, améliorer encore les choses ?

Le vote du 15 janvier prolonge la période d'incertitude qui s'est ouverte il y a deux ans lorsque les Britanniques ont voté en faveur du Brexit. Certes, la France se prépare à faire face aux situations les plus urgentes si aucune solution n'est trouvée d'ici au 29 mars prochain. La Commission européenne prépare de son côté quatorze mesures visant à atténuer les conséquences immédiates d'un Brexit sans accord. En effet, le rejet par le Parlement britannique de l'accord passé entre le Gouvernement britannique et l'Union européenne remet en cause les dispositions négociées depuis septembre 2016. Cela aura notamment des conséquences sur le statut, les droits et la liberté de circuler des ressortissants français résidant au Royaume-Uni. L'accord négocié prévoyait le maintien des droits des ressortissants européens jusqu'à la fin de la période de transition, fixée au 31 décembre 2020. Cela assurait à nos concitoyens résidant au Royaume-Uni la possibilité d'y vivre, d'y travailler ou d'y étudier dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Cet accord leur donnait le droit de continuer à résider au Royaume-Uni, à condition de faire la demande d'un statut de résident permanent avant le 30 juin 2021.

qui les concerne, de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne au bout de huit ans. Le Sénat avait alors également demandé qu'un protocole distinct de l'accord de retrait soit établi pour garantir les droits des ressortissants européens- dont français -en cas d'échec des négociations. À ce jour, il n'existe toujours pas. La Commission européenne, tout comme le projet de loi français, prévoit la garantie d'un certain nombre de droits pour les ressortissants britanniques résidant sur le continent après le 29 mars, mais sous réserve de réciprocité.

si le Brexit ne veut rien dire, alors le Brexit ne doit pas être. Cependant, le Brexit sans accord reste une option sur la table.

Chaque jour, des associations de défense qui les représentent, comme The3million, In Limbo Project ou encore British in Europe, se font l'écho d'une grande désespérance, d'une xénophobie ambiante et de drames humains. la situation de ces familles qui risquent de voler en éclats, car certains de leurs membres ne seront plus les bienvenus au Royaume-Uni, du fait de l'application de nouveaux critères liés à la nationalité ou aux revenus. Ce Brexit a déjà un coût humain déplorable.

pensez-vous que cela puisse être encore envisageable ?

un nouveau projet lundi prochain. Effectivement, les parlementaires britanniques réfléchissent à un certain nombre d'options. Vous vous souvenez sans doute

Nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer le début, mais nous pouvons commencer où nous sommes et changer la fin. » C'est par cette citation de l'écrivain britannique C.S. Lewis que le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans a conclu hier matin son intervention devant le Parlement européen.

et des préoccupations liées non seulement au retrait du Royaume-Uni, mais également à la fragilisation de l'Union européenne et à l'instabilité actuelle du monde. Mais il est une réalité qu'aucun scénario ne peut changer : avec ou sans accord de sortie d'ici au 29 mars prochain, le Royaume-Uni ne sera jamais et ne pourra jamais être,, considéré comme un pays tiers. Le Royaume-Uni est la sixième puissance économique mondiale ; derrière l'Allemagne et la France, il est le troisième pays européen en termes de population, et il représente le premier excédent commercial de la France au sein de l'Union européenne. L'accord de sortie comme la déclaration politique sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne portent sur le cadre juridique, réglementaire, institutionnel et financier, et il ne sera pas définitivement documenté, dans tous les cas, d'ici au printemps, en ce qui concerne les relations qui s'ouvriront après la période de transition, d'ici à 2020 ou à 2022. La France et le Royaume-Uni ont ouvert une nouvelle ère dans leurs relations matière de défense, depuis les traités de Lancaster House de 2010, puis le sommet d'Amiens de 2016. Dès lors, le retrait britannique de l'Union européenne investit la France d'une responsabilité particulière, à l'égard tant du Royaume-Uni que de l'Union européenne et du monde.

de l'Union européenne. Aussi, madame la ministre, le Gouvernement envisage-t-il la mise en place d'une stratégie claire de promotion et d'enseignement du français dans le cadre de l'Union européenne et de ses institutions, voire au-delà ? La parole est

Même en cas de retrait sans accord, nous en viendrons à négocier un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni, car nombre de liens,

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret. Le vote du Parlement britannique nous place dans une situation inédite et redoutée. Il ne doit pas nous empêcher de continuer à nous préparer à toutes les options, voire à saisir de nouvelles opportunités. Je rentre d'une mission en Irlande. Mes interlocuteurs et notre ambassadeur m'ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'impact négatif du Brexit sur l'activité économique, mais ils ont aussi souligné l'occasion qu'il représente de renforcer notre relation bilatérale. Ils pensent notamment à l'ouverture de nouvelles routes maritimes entre l'Irlande et la France. Or, comme l'indique la résolution adoptée par le Sénat en novembre dernier sur la question des corridors maritimes -je salue à cet égard le travail des corapporteurs, Didier Marie, Pascal Allizard et Jean-François Rapin la Commission européenne n'a pas pris en compte les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni, notamment dans l'hypothèse d'une sortie sans accord, sur le fret maritime entre la République d'Irlande et le continent européen. Aucune étude solide n'a été réalisée sur une réorientation des flux de marchandises à destination de la République d'Irlande. Pourtant, ils transitent aujourd'hui à hauteur de 80 % par le Royaume-Uni, les exportations irlandaises représentent 42 % du PIB. Tout nous incite donc aujourd'hui à entamer des négociations avec la République d'Irlande afin d'ouvrir de nouvelles routes maritimes et éviter qu'elle ne soit victime du chaos annoncé en matière douanière. À l'occasion des travaux d'aménagement en cours des ports français, nous pourrions ainsi envisager la mise en place de couloirs dédiés aux camions de fret en direction ou en provenance d'Irlande. Cette question de l'aménagement est aujourd'hui complexe et urgente ; il est nécessaire d'y dédier fonds et personnels supplémentaires. Nous savons que vous avez déjà établi un premier dialogue avec le ministre irlandais des affaires étrangères et du commerce en octobre dernier. Qu'est-il ressorti de ces premiers échanges ? Soutiendrons-nous la demande d'une aide financière de l'Union européenne en cas de Brexit sans accord ? Entendez-vous donner suite à notre résolution, qui vous invite à engager sans tarder une réflexion sur les flux commerciaux entre l'Irlande et le continent ? La parole est à Mme la ministre.

en rappelant par ailleurs que les capacités militaires britanniques représentent entre 25 % et 30 % des capacités totales de l'Union européenne. Peut-on raisonnablement s'en passer ? Tout le monde convient que le degré de coopération entre Bruxelles et Londres sur les questions de sécurité et de défense doit être le plus élevé possible. Oui, mais comment faire, concrètement ? ? Les Britanniques proposent, dans le Livre blanc sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne de juillet 2018- c'est le point 68-et la note technique du 24 mai 2018, de participer à des réunions informelles du Comité politique et de sécurité, le COPS, et du Conseil des affaires étrangères, le CAE. Les Britanniques proposent donc de participer à des réunions informelles des organes décisionnels

que se passera-t-il après le Brexit ? Cette position ferme sera-t-elle maintenue ? Enfin, quelle sera la future relation entre le Royaume-Uni et l'Europe de la défense ? La parole

en matière de défense. J'oserai même dire que s'il est un domaine où l'Europe a réussi à avancer ces derniers mois du fait du retrait britannique, c'est vraisemblablement celui de l'Europe de la défense, à laquelle les Britanniques ont toujours été résolument hostiles. Aujourd'hui, au moment où ils quittent l'Union européenne, ils se prennent d'une affection nouvelle pour cette Europe de la défense, parce qu'elle voit le jour. Ainsi, ils ont demandé à participer

Eh bien ce n'est pas possible : en bon anglais,. En effet, l'un des principes sur lesquels nous avons fondé nos directives de négociation est la préservation de l'autonomie de décision de l'Union européenne, un principe auquel les Britanniques eux-mêmes étaient fortement attachés

de travailler avec eux à l'évaluation de la menace, à la planification commune, à la création d'une culture stratégique commune entre pays européens, au sens géographique du terme, capables et volontaires, y compris le Royaume-Uni.

Gaulle le 17 juillet 1961. « Ou bien c'est l'Europe qui défendra elle-même son territoire, ou bien il n'y aura pas, pour l'Europe, de défense qui tienne. « Il y a l'OTAN. Qu'est-ce que l'OTAN ? C'est la somme des Américains, de l'Europe et de quelques accessoires. Mais ce n'est pas la défense de l'Europe par l'Europe, c'est la défense de l'Europe par les Américains. Il faut une autre OTAN.

aux Britanniques, dans un contexte européen difficile, où la montée des populismes et le rejet global de l'Union européenne dominent.

Comment sortir de cette situation sans pénaliser durablement la qualité de nos relations avec les Britanniques, tout en préservant la cohésion des vingt-sept États membres ?

des États membres de l'Union européenne ? C'est précisément tout l'objet du travail d'orfèvre mené par Michel Barnier, qui a conduit à l'accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni.

particulières que sont les ports et le tunnel sous la Manche. Une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord aura un impact considérable sur les flux de marchandises et de personnes.

sont au bord de l'épuisement, comme l'a souligné très récemment notre collègue François Grosdidier dans un rapport sur le malaise des forces de sécurité intérieure.

afin de séparer de la manière la plus claire possible les camions en provenance du Royaume-Uni, qui devront faire l'objet d'un certain nombre de contrôles, et les camions à destination du Royaume-Uni, qui sont, nous le savons, un point de fixation pour les trafics De ce point de vue, la coopération bilatérale franco-britannique est étroite en matière lutte contre les trafiquants d'êtres humains. Cette coopération, qui fonctionne à plein, a vocation à se poursuivre et à se développer encore.

demande. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le scénario tant redouté est donc advenu. La Grande-Bretagne et l'Union européenne entrent en territoire inconnu. La tonalité générale de notre débat témoigne bien d'un profond désarroi, même si nous pouvions nous attendre à cette issue. L'Union européenne et ses États membres, dont la France, ont préparé ces derniers mois des dispositions d'urgence pour faire face à une telle éventualité. Nous espérions tous, en notre for intérieur, que ces précautions indispensables n'auraient pas à s'appliquer. Nous péchions sans doute par excès d'optimisme. Aussi précises soient-elles, ces mesures n'empêcheront cependant pas l'impact désastreux que la décision du Parlement britannique aura pour les deux parties. On sait que plusieurs secteurs économiques seront directement touchés par la sortie du Royaume-Uni. L'industrie française est concernée au premier chef et devra relever plusieurs défi logistique, d'abord, avec l'augmentation du délai des formalités douanières à la frontière, qui provoquera des goulets d'étranglement. Un défi des tarifs douaniers, ensuite : en l'absence d'accord de libre-échange, le Royaume-Uni pourrait instaurer des tarifs douaniers élevés, par exemple dans le secteur automobile, comme autorisé par l'Organisation mondiale du commerce. Cette organisation, bien qu'elle soit chancelante en ce moment, va en effet devenir, pour la Grande-Bretagne, le cadre naturel des négociations commerciales sur les tarifs douaniers et les barrières non tarifaires, dans l'hypothèse d'un Brexit « dur ». Que dire, enfin, sur l'avenir de la pêche européenne, et en particulier de la pêche française ? Une fermeture des eaux britanniques induirait une perte de revenus, pour la flotte européenne, de l'ordre de 50 %. Certes, le choix de ne pas rester dans l'Union européenne n'implique pas une rupture totale de nos relations avec le Royaume-Uni.

Comment trouver désormais une solution acceptable par tous en ce qui concerne la frontière physique entre l'Irlande et l'Ulster, qui devient désormais « la » frontière terrestre entre l'Union et le Royaume-Uni, alors même que, depuis 1998, l'Union est,

nul n'est parvenu, malgré quelques tentatives, à en ébranler la solidité. J'y vois deux raisons essentielles. La première est la qualité du négociateur en chef Michel Barnier. Il faut lui faire crédit d'avoir contribué, avec beaucoup de patience et de talent, à créer et, surtout, à maintenir cette solidarité politique des Vingt-Sept, qui était loin d'être acquise de prime abord. La seconde raison est que la lucidité, l'honnêteté politique et la clarté des principes de base de la négociation auront été, durant ces mois, beaucoup plus présentes du côté des Vingt-Sept que de l'autre. Ce sont là des qualités dont on crédite trop peu souvent l'Union européenne et ses institutions ; c'est l'occasion de le faire. Le résultat du vote de mardi est un revers pour tout le monde : pour les Britanniques d'abord, mais aussi pour l'Union. C'est aux Britanniques désormais et à eux seuls, en particulier à leur Parlement, qu'il revient d'inventer un « plan B » pour baliser le chemin qui mène au 29 mars.

Au-delà de cet écueil, il reviendra aux Vingt-Sept, à la Commission européenne et au futur Parlement européen de continuer et d'amplifier le travail de refondation de l'Union. Le Conseil européen de Sibiu, en mai, sera une première étape importante. Enfin, comme son intitulé l'indique, notre groupe sénatorial de suivi sur le retrait du Royaume-Uni et la refondation de l'Union européenne, que Christian Cambon et moi-même avons l'honneur de présider, n'a jamais dissocié les deux enjeux. Il poursuivra ses travaux

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Brexit, décidé au Royaume-Uni, aura des conséquences dans toute l'Europe. Ce divorce est déjà douloureux. Il le sera encore davantage dans les prochains mois lorsqu'il sera effectif et qu'il faudra le mettre en oeuvre. Il est donc nécessaire de s'y préparer. C'est ce que le Gouvernement nous propose de faire par voie d'ordonnances avec ce projet de loi d'habilitation, sur lequel la commission mixte paritaire a trouvé un accord. Le vote négatif du Parlement britannique du 15 janvier réactualise l'hypothèse d'un Brexit « dur », sans accord, que nous redoutions depuis le début du processus. Les dirigeants européens ont rappelé, à juste titre, que l'accord signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne le 25 novembre 2018 n'était pas négociable. Cet accord est en effet le seul possible, car il ménage une clause de sauvegarde sur la frontière irlandaise et préserve les intérêts essentiels de l'Union Nous sommes reconnaissants à Michel Barnier d'être parvenu à élaborer ce texte en maintenant un front uni des Vingt-Sept, ce qui n'était pas évident au départ ! Certains, aujourd'hui, espèrent que le Brexit n'ait finalement pas lieu. Ne rêvons pas ! Nous avons surtout le devoir d'intensifier notre préparation aux conséquences juridiques, économiques et sociales d'un Brexit « dur ». Les citoyens, les entreprises, ne sont pas encore tous et toutes conscients de ce que ce scénario implique. Le Brexit « dur » est un divorce non ordonné et sans phase de transition, revenant à effacer brusquement quarante-cinq ans d'acquis européen. Nous sommes inquiets des conséquences économiques de cette situation sur le secteur agroalimentaire, sur la pêche, ainsi que sur de nombreux secteurs industriels, notamment celui de l'automobile. les Britanniques craignent des pénuries, notamment dans le secteur du médicament. Les défis logistiques sont considérables. Le ministère britannique des transports estime, par exemple, que l'axe Douvres-Calais pourrait ne fonctionner qu'à seulement 13 % de ses capacités pendant les six premiers mois suivant le Brexit. Notre autre préoccupation essentielle, ce sont bien sûr les droits des citoyens. L'accord du 25 novembre 2018 apportait un certain nombre de garanties qui seraient remises en cause faute de ratification. Les citoyens européens du Royaume-Uni et les citoyens britanniques résidant dans l'Union européenne, qui n'ont d'ailleurs pas eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre du référendum sur le Brexit, sont aujourd'hui dans l'incertitude la plus totale.

instants -, ces mesures ont vocation à être temporaires, dans l'attente d'une solution globale ou d'un accord bilatéral avec le Royaume-Uni. La Constitution a le mérite de permettre à la France d'agir vite lorsque c'est nécessaire, mais cette possibilité est encadrée : il ne s'agit pas de donner un blanc-seing au Gouvernement. C'est pourquoi le Sénat a précisé l'habilitation, tant dans ses finalités que dans ses champs d'intervention, non pas pour fragiliser l'action du Gouvernement, mais, au contraire, pour la consolider juridiquement, car des recours ne sont pas à exclure. Nous avons notamment précisé le régime applicable aux travaux urgents rendus nécessaires par le rétablissement des contrôles aux frontières. Le Sénat a également souhaité renforcer l'attractivité du territoire français pour les Britanniques appelés à exercer une activité en France après le Brexit et faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues au Royaume-Uni après le Brexit. L'Assemblée nationale a conservé la structure et la philosophie générale du texte adopté par le Sénat. Je remercie d'ailleurs le rapporteur Alexandre Holroyd, avec lequel nous avons noué un dialogue franc et constructif. Ainsi, nous avons eu le souci commun de préserver l'attractivité de la France, pour les entreprises britanniques qui souhaiteraient s'y redéployer. Nous nous sommes également accordés sur une disposition innovante relative au contrôle parlementaire de la préparation et de la mise en oeuvre des ordonnances. Notre groupe de suivi du Brexit, présidé par Jean Bizet et Christian Cambon, que je tiens à saluer, disposera ainsi des moyens de poursuivre l'action menée depuis près de deux ans et demi. Mes chers collègues, en définitive, nous avons pu travailler avec le rapporteur de l'Assemblée nationale à un compromis qui me paraît satisfaisant. Ainsi, la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun, que je vous propose aujourd'hui d'adopter. Toutefois, madame la ministre, beaucoup reste à faire. La balle est maintenant dans votre camp. Le Brexit est un changement structurel, qui aura des impacts à long terme et qui constitue, dans l'immédiat, un facteur d'incertitude supplémentaire, alors que la France

nous avons largement eu l'occasion de le dire au cours du débat qui a précédé : le rejet, à une très large majorité- 230 voix d'écart -, de la ratification du projet d'accord de retrait par la Chambre des communes, le 15 janvier dernier, accroît les incertitudes quant aux conditions du retrait britannique. Il aggrave fortement les risques de perturbations résultant du retrait et la probabilité d'un Brexit sans accord, qui risquerait d'affecter durement, si nous n'agissions pas, les citoyens, les acteurs économiques et l'ensemble des parties prenantes.

nationale, le Premier ministre a demandé, dès le mois d'avril 2018, à l'ensemble des ministères d'identifier les conséquences d'une absence d'accord et les mesures à prendre. Ce travail s'est notamment traduit dans un projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires en cas d'absence d'accord. Nous en avons discuté ici même,

cinq ordonnances seront bientôt prêtes à être présentées au conseil des ministres- la première d'entre elles sera examinée dès la semaine prochaine. Elles couvriront trois domaines, que je tiens à rappeler. Le premier est la situation des ressortissants français qui vivent au Royaume-Uni et qui reviendraient en France et, de manière plus générale, les intérêts français, notamment dans le domaine de la défense ou en matière financière. Le deuxième est la situation des Britanniques en France, qu'il s'agisse, par exemple, des droits d'entrée et de séjour, de l'emploi ou des prestations sociales, étant entendu que ces mesures seront prises dans un esprit de réciprocité. troisième et dernier est la circulation des personnes et des marchandises. Même en cas d'accord, il conviendra de réaliser les travaux de construction ou d'aménagement de locaux, installations, infrastructures portuaires, ferroviaires, aéroportuaires et routières qui seront requis par le rétablissement des contrôles de marchandises et de passagers à destination et en provenance du Royaume-Uni. Dans ces trois domaines, il s'agit seulement d'assurer les éléments de continuité indispensables, de façon temporaire, avant l'entrée en vigueur, soit d'un accord de retrait, soit directement d'accords européens et nationaux encadrant les relations futures. les travaux menés avec le Sénat comme avec l'Assemblée nationale au titre de ce projet de loi ont permis des avancées rapides et substantielles. L'adoption et la promulgation de ce texte avant la fin du mois de janvier permettront ainsi de placer la France, avec l'Allemagne, parmi les États membres les plus avancés, au sein des 27, dans la préparation à une sortie sans accord. Le projet de loi sur lequel vous avez travaillé constitue une référence pour plusieurs de nos partenaires européens. Je tiens donc à remercier le Sénat d'avoir pris toute la mesure de l'urgence de la situation à laquelle nous devons faire face, et d'avoir considéré, au vu de son caractère inédit et de l'importance des enjeux, qu'il pouvait accepter l'habilitation sollicitée. Je tiens également à vous remercier des discussions que nous des discussions que nous avons eues au cours de l'examen de ce projet de loi d'habilitation, ainsi que de vos contributions. Je salue notamment le travail relatif à la structure de ce projet de loi, puisque vous souhaitiez mieux faire ressortir la finalité des ordonnances, ainsi que les précisions utiles que vous avez apportées quant à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Au-delà Au-delà de ce projet de loi d'habilitation et des ordonnances qui seront prochainement adoptées sur ce fondement, le Gouvernement ne ménage aucun effort pour limiter autant que possible les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni sans accord.

qu'il s'agisse de personnels, d'équipements ou de la construction d'infrastructures. J'ai ensuite pris part, aux côtés du Premier ministre, à un déjeuner avec les présidents de région

dossier. Des mesures d'information et de communication ont également été prises, en particulier à travers la création d'un site internet interministériel unique d'information dédié au Brexit. Ce site vise à donner des informations générales et à répondre aux questions que se posent les particuliers et les entreprises. Nous nous préparons à une communication beaucoup plus active et vigoureuse dans ce domaine, mais- je n'en doute pas -le vote du 15 janvier dernier aura pour effet de rendre nos concitoyens et nos entreprises plus sensibles aux risques d'une absence d'accord et à la nécessité de s'y préparer. Enfin, je vous

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi aujourd'hui soumis à notre approbation est le fruit d'une commission mixte

mixte paritaire du 18 décembre dernier : l'urgence de préparer au mieux notre pays aux conséquences du Brexit justifiait le pragmatisme et la flexibilité dont le Parlement a su faire preuve en cette occasion. madame la ministre, ce n'est pas rien pour des parlementaires, notamment dans un régime comme le nôtre, marqué par la prééminence de l'exécutif, d'accepter le recours aux ordonnances en lieu et place de la production ordinaire de la loi. Les négociations conduites par nos deux rapporteurs spéciaux ont heureusement permis, en contrepartie de notre acceptation de légiférer par ordonnances, de renforcer le rôle du Parlement dans l'élaboration, le contrôle et l'évaluation de ces mêmes ordonnances. Il s'agit là d'une très bonne chose.

il démontre, s'il le fallait encore, que l'intelligence et le pragmatisme de notre représentation nationale, au-delà de ses habituels clivages politiques, ont de quoi faire pâlir de jalousie certains de nos homologues d'outre-Manche étant, les raisons de nous réjouir s'arrêtent malheureusement là ; car si la Première ministre britannique est parvenue hier soir, et de justesse, à sauver sa place malgré la motion de défiance présentée

qu'un Brexit dur aura pour l'économie européenne en général, et pour l'économie française en particulier. Ces derniers mois, certains d'entre nous se sont parfois enthousiasmés des possibles retombées positives du Brexit pour notre économie, notamment pour la place financière de Paris. Ils oubliaient un peu vite que c'est avec son voisin d'outre-Manche que notre pays jouit de son plus fort excédent commercial ... Notre secteur agroalimentaire a

Ce livre collectif décrivait avec sévérité les atermoiements de la Grande-Bretagne face aux changements en Europe et dans le monde, son attachement à un Commonwealth périmé, que la décolonisation rendait obsolète, son hésitation à adhérer au Marché commun et sa nostalgie d'une grandeur passée qui privait la société britannique de tout dynamisme.

: « Voilà comment l'ADN démocratique d'un très grand pays européen a été génétiquement modifié par une bande de voyous populistes, j'ai nommé principalement Boris Johnson et Nigel Farage, des hommes qui ont prospéré sur le mensonge à des fins purement politiciennes, et dont le comportement,

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce débat sur la demande d'habilitation du Gouvernement à prendre des mesures de préparation au retrait britannique illustre, comme nous l'avons souligné lors de la première lecture, la crise que traversent aujourd'hui l'Union européenne et le projet européen Nous l'avons souligné : cette crise est inédite par sa gravité et son ampleur, car elle dépasse le cas britannique. L'Union européenne n'est plus, aux yeux de tous, à même de faire la richesse des nations ou d'assurer la prospérité des peuples.

Ainsi, après le vote d'un amendement à la loi de finances qui a fixé des limites au pouvoir du Gouvernement de modifier, à la suite du Brexit, la réglementation relative aux taxations indirectes, de nombreux observateurs de la vie institutionnelle britannique

L'exécutif britannique a donc trois jours pour présenter un nouvel accord au Parlement, au risque de laisser la possibilité à ce même Parlement de définir les conditions du Brexit, si le Gouvernement n'y parvenait pas.

Le Parlement est un véritable contre-pouvoir à l'exécutif, et les parlementaires de la majorité ne sont pas de simples godillots. C'est aussi cela, une véritable démocratie représentative.

Cette dernière a pourtant fait du bon travail et n'a pas cherché à enquiquiner le Gouvernement en le mettant en difficulté. Elle a, au contraire, tenté très sincèrement d'aider en tenant compte de la situation des Britanniques, y compris après le Brexit, qu'il y ait ou non accord. » Nous l'avions déjà souligné au sujet de ce projet d'habilitation : même si l'urgence est réelle, le Gouvernement demande des pouvoirs dérogatoires à nos yeux trop étendus, qu'il s'agisse de l'urbanisme, de l'aménagement, du respect du droit de l'environnement ou des règles de la commande publique. D'ailleurs, nous l'avons souligné lors des débats, la question des aménagements nécessaires afin d'assurer le contrôle des marchandises et des passagers en provenance et à destination du Royaume-Uni n'est pas nouvelle, tout comme la faiblesse de nos ports, par manque de vision claire et, surtout, d'investissements. en première urgence, dès le début du quinquennat, qu'il aurait fallu construire des bureaux de douane et recruter les agents nécessaires à l'anticipation de cet événement historique qu'est le Brexit. Toutefois, la finalité des ordonnances telle que précisée par le Sénat a été préservée, et l'information du Parlement a été renforcée. Aussi, comme en première lecture, nous nous abstiendrons sur ce texte, malgré notre opposition de principe aux demandes d'habilitation, aussi le fait que la situation d'urgence est pour partie le fait du Gouvernement, qui aurait dû anticiper l'hypothèse d'une sortie britannique sans accord ; il a d'ailleurs montré sa capacité à le faire en matière fiscale ou financière, lorsqu'il s'agissait de « renforcer » l'attractivité de la place financière de Paris. nous abstiendrons, car le sort des ressortissants britanniques installés en France et des Français installés au Royaume-Uni ne peut souffrir d'incertitudes ; le projet d'habilitation permet

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, de l'Entente cordiale nos jours, les relations entre le Royaume-Uni et notre pays sont le fruit d'une longue construction qui a tenu bon malgré les soubresauts de l'histoire, particulièrement lorsque cette dernière s'est montrée sous son jour le plus tragique, lors de la Seconde Guerre mondiale. Nos deux pays sont liés, et ils le resteront au-delà de la volonté des électeurs britanniques de sortir de l'Union européenne. Ils sont liés parce qu'ils sont voisins et à peine séparés par une bande de mer large

nos regrets, nous ne pouvons qu'accompagner du mieux possible la décision de sortie de l'Union européenne. C'est dans cet état d'esprit que nous avons abordé l'examen de ce projet de loi, et c'est dans cet esprit que nous poursuivrons notre travail. Mais, depuis l'annonce des résultats du référendum, la situation a pris une drôle de tournure. Le dernier soubresaut est survenu avec le vote de la Chambre de communes, ce mardi 15 janvier, qui s'est soldé par le rejet de l'accord sur le Brexit. sur le Brexit. Aucun doute n'a été levé par le Royaume-Uni ; pis encore, de nombreuses incertitudes viennent aggraver une situation déjà hasardeuse. Ce projet de loi doit permettre de préparer l'éventualité d'un Brexit sans accord. Mais, en tout état de cause, il ne permettra que de gérer cette urgence, et toutes les incertitudes ne pourront être levées. De très nombreux points d'inquiétude subsistent, d'autant que, malgré ces mesures pour lesquelles le Gouvernement nous demande notre habilitation, malgré les efforts consentis, nous serons difficilement prêts, en cas de Brexit, le 29 mars 2019. 2019. Dans tous les cas, le degré d'impréparation du Royaume-Uni ne manquera pas d'avoir de lourdes conséquences. Au rang de nos inquiétudes se trouve notamment la gestion des espaces frontaliers qui voient transiter, à titre d'exemple, plus de 5,2 millions de camions chaque année.

sur l'organisation et les activités de nos ports maritimes. Ces derniers méritent autant son attention que les ports hollandais et belges. Je pense notamment aux ports de Cherbourg et du Havre, les équipements et les personnels doivent certes être renforcés, mais dont le savoir-faire n'est plus à démontrer pour absorber les flux venus d'Irlande dans les meilleures conditions possible. Je réitère également, au nom de mon groupe, les propos tenus par mon ami Didier Marie : à nos yeux, notre travail de parlementaires est d'accompagner le Gouvernement, en lui donnant les moyens d'agir avec flexibilité et réactivité, notamment par l'outil des ordonnances. Mais cette méthode doit engager le Gouvernement à garantir la plus grande transparence, en permettant au Parlement d'exercer pleinement ses capacités de contrôle. Sur ce dernier point, nous serons inflexibles. Le Parlement doit pouvoir contrôler avec régularité et précision toutes les actions du Gouvernement dans le processus de sortie de l'Union européenne qu'a engagé le Royaume-Uni.

C'est pourquoi nous avons apprécié la rédaction proposée par l'Assemblée nationale au premier alinéa de l'article 4 ; elle exprime le souci de garantir un véritable contrôle parlementaire, aussi bien sur la préparation des ordonnances que sur la mise en oeuvre des mesures décidées dans le cadre de cette procédure. texte confère une large marge d'action au Gouvernement pour prendre des mesures dérogatoires en matière d'aménagement, d'urbanisme et de règles relatives aux commandes publiques.

nous voyons les conséquences d'un référendum dans une démocratie considérée, à juste titre, comme exemplaire depuis des siècles.

Nos deux pays ont construit un tunnel, surtout payé, d'ailleurs, par les petits actionnaires français, par lequel nous espérions arrimer la Grande-Bretagne au continent, dans le respect de sa différence.

Ce qui se passe est extrêmement grave. Madame la ministre, vous avez beaucoup travaillé en amont ; le Parlement aussi, tout particulièrement le Sénat. Et, par les temps qui courent, il m'est agréable de rappeler l'utilité du Sénat

tant que ministre, j'ai dû y recourir, mais vous savez que je l'ai fait avec douceur, et en les réduisant au minimum. Cela étant, en la matière, il était pratiquement impossible de faire autrement.

sous le précédent quinquennat, lors des premiers débats sur le Brexit, combien il était important aussi de rappeler les liens que nous avons avec la Grande-Bretagne et de ne rien faire, de notre côté, qui puisse accentuer la fracture, tout en étant très fermes sur les conditions de négociation. Il ne faut jamais oublier que des des Grands-Bretons, comme nous disons, ont beaucoup fait pour notre pays dans les heures les plus sombres. Je ne puis ainsi jamais parler du Brexit sans avoir une pensée pour Winston Churchill, qui a tant fait pour

encore davantage d'incertitudes sur les conditions de la sortie de ce pays de l'Union européenne. Le scénario du étant de plus en plus probable, cela justifie plus que jamais la prise de mesures d'urgence, donc l'adoption de ce texte. Malgré le flou qui entoure cette affaire depuis son commencement, il est certain que les effets attendus d'un Brexit sans accord seront probablement graves pour l'économie, tant britannique que française et européenne. Ainsi, dans mon département, le Nord, mais aussi dans le Pas-de-Calais et dans les territoires qui de très nombreuses entreprises commercent quotidiennement avec le Royaume-Uni et sont dépendantes du principe de libre circulation qui est aujourd'hui remis en cause. d'ailleurs pas certain- c'est un euphémisme ! -que les entreprises aient pris la juste mesure des conséquences et qu'elles soient toutes prêtes. Il ressort également que les infrastructures routières et portuaires ne sont pas adaptées aux longues files d'attente qu'entraînera nécessairement la remise en place de contrôles douaniers et sanitaires. Or la fluidité du trafic transmanche est essentielle pour l'activité de ces entreprises, et il en va de même pour des milliers d'entreprises ailleurs en France, tout comme chez nos voisins continentaux. Nos collectivités et nos entreprises ne pourront pas seules faire face à un changement aussi radical et brutal. L'État et les autorités européennes doivent les accompagner et les protéger. Le Brexit n'affectera pas seulement notre économie : il impactera aussi les droits de nos citoyens établis outre-Manche, la fonction publique, les étudiants en mobilité, et bien d'autres domaines encore. Le projet de loi a justement pour objet de répondre à ces enjeux, et le Gouvernement entend pour cela procéder selon un principe général de réciprocité. Si cette approche est légitime et indispensable, l'absence d'indications de la part de nos partenaires britanniques sur leurs intentions limite nécessairement sa mise en oeuvre. En clair, le problème est que ni le Parlement britannique ni l'opinion britannique ne savent réellement ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs une leçon sur les dangers des consultations populaires improvisées : il est plus facile de construire des majorités contre que des majorités pour. C'est à méditer, alors même que le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, surgit dans le débat politique français. David Cameron a voulu jouer au plus malin, et tel le rat avec l'huître dans les fables de La Fontaine, « tel est pris qui croyait prendre ». Dans la presse de ce matin, il a dit qu'il ne regrettait rien. diable, un peu d'humilité ferait du bien ! Je crois que David Cameron, tout comme le référendum en Angleterre, est hors-jeu pour longtemps, voire pour toujours. Tant mieux ! N'est pas Churchill qui veut de cette situation de confusion, je veux saluer le travail constructif des deux assemblées. Le Parlement n'est évidemment, cela a été dit, que rarement favorable au recours aux ordonnances. Nous reconnaissons cependant que cette méthode est la plus adaptée pour faire face à l'urgence de la situation. Je pense notamment aux procédures d'urgence en matière d'urbanisme et à beaucoup d'autres encore. La commission mixte paritaire a abouti à un texte équilibré, à même de permettre au Gouvernement de remplir pleinement ses objectifs pour limiter l'impact du tout

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « les bons Européens sont ceux qui savent identifier les difficultés, essaient de les résoudre et ne se laissent jamais décourager Il nous revient plus que jamais de suivre cette phrase de Paul-Henri Spaak et de ne pas nous décourager face à la décision radicale prise mardi par la Chambre des communes britannique. Le Royaume-Uni semble en effet avoir décidé de mettre fin de façon désordonnée à ses quarante-six ans d'appartenance à l'Union européenne, en rejetant un texte négocié durant plus de dix-sept mois ; je tiens, à cet égard, à saluer l'excellent travail mené par Michel Barnier. Ce rejet plonge le Royaume-Uni et l'Union européenne dans un état d'incertitude inédit. Pourtant, en décembre dernier, Theresa May a réussi à repousser le vote dans l'espoir de parvenir à un accord avec les députés ou d'arracher une concession à Bruxelles. Échec des deux côtés. Or, en parallèle, l'horloge continue de tourner, la date du Brexit se rapproche : soixante-dix jours pour éviter de rompre dans le chaos et l'urgence. Les semaines à venir s'annoncent, à la fois, décisives et terriblement incertaines. À l'heure du premier bilan, il est difficile d'évaluer la performance de Theresa May. Force est de constater que, en dépit d'élections anticipées catastrophiques, des démissions en série, des confrontations défavorables à Bruxelles, des revirements récurrents et des fausses informations répandues sur les réseaux sociaux, Theresa May a su faire preuve d'une capacité de résilience peu commune. On ne peut que l'admirer pour cela. Comment ne pas en vouloir à cette classe politique britannique, première responsable de cette faillite collective, à commencer par le parti conservateur, qui risque de précipiter tout le Royaume-Uni dans un Brexit sans accord dont personne ne voulait Et que dire de cette coalition baroque regroupant les eurosceptiques et européistes irréductibles, les Écossais indépendantistes et les Nord-Irlandais unionistes, des conservateurs et des travaillistes, réunis pour s'opposer à un accord pour des raisons bien différentes les unes des autres ? Dès lors, que faire ? Plusieurs hypothèses sont sur la table : renégociation de l'accord, nouveau référendum, élections anticipées,, Brexit sous conditions, motion de défiance ... Certains évoquent même un report de la date du 29 mars, avec des conséquences ubuesques sur les élections européennes du 26 mai. Il est consternant de constater que l'Europe est totalement impuissante et dépendante de la dynamique politique anglaise, alors même que les Européens ont multiplié les efforts et les signaux, y compris pour rassurer les Anglais sur le irlandais. Il convient de ne pas oublier que ce projet d'accord, froidement rejeté par le Royaume-Uni, s'inscrit à bien des égards dans une perspective plus large, celle de la construction d'une relation future entre les Européens et les Britanniques. La France devra oeuvrer avec ses partenaires européens, en maintenant l'unité et la solidarité des Vingt-Sept, pour trouver rapidement des solutions communes et pérennes. Le Royaume-Uni est et doit rester, d'une façon ou d'une autre, un partenaire de la France et de l'Europe. Nous devons aller de l'avant, assurer cette continuité, mais aussi penser à l'avenir de l'Union européenne à vingt-sept, ainsi qu'à nos concitoyens, et veiller à répondre au mieux à leurs attentes. De plus en plus d'hommes et de femmes sur notre continent ont le sentiment de ne pas être écoutés par une Europe qui se ferait sans eux. Les élections européennes de mai prochain, perturbées par le Brexit, ne doivent pas devenir une occasion ratée de faire vivre notre démocratie européenne. Pour cela, il faut tout d'abord sécuriser les relations avec le Royaume-Uni, en prenant rapidement les mesures d'urgence nécessaires. Déjà, les États membres commencent à prendre des mesures pour éviter tout vide juridique en cas de la la Commission européenne a sorti en décembre un plan d'action d'urgence comprenant quatorze mesures pour éviter que ce scénario catastrophe ne heurte trop ses intérêts ses intérêts « vitaux », ceux de ses 450 millions de citoyens et de ses dizaines de milliers d'entreprises. Mais, nous le savons, c'est loin d'être suffisant. Ce projet de loi, qui prévoit la mise en oeuvre d'ordonnances en France, n'est sûrement pas la panacée. Toutefois, il permet de répondre dans l'urgence à un et de préserver les intérêts des citoyens et des entreprises. Il permettra d'éviter que les 150 000 ressortissants anglais en France n'aient plus le droit de séjourner, que des avions ne soient cloués au sol ou que des médicaments ne puissent plus arriver jusqu'aux Britanniques, et de la même façon jusqu'en France, aggravant ainsi de part et d'autre le problème de la pénurie de médicaments. Madame la ministre, les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires espèrent que le Gouvernement n'aura pas à prendre ces ordonnances. Cela signifierait l'échec des négociations

mauvais Nous voterons, bien entendu, en faveur de ce texte tel qu'il a été amendé par la commission mixte paritaire. Bizet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises lors de l'examen de ce projet de loi en première lecture, les parlementaires apprécient généralement peu le recours aux ordonnances. À cette occasion, nous avions néanmoins largement estimé sur ces travées que la grande incertitude sur le devenir de l'accord de retrait entre l'Union et le Royaume-Uni permettait de justifier cette solution, en réalité la seule possible pour permettre au Gouvernement d'adopter, dans l'urgence, les mesures qui s'imposent afin de limiter les effets néfastes du Brexit, tout particulièrement en cas d'absence d'accord. Justement, le rejet mardi soir par la Chambre des communes de l'accord de retrait et de la déclaration politique sur les futures relations euro-britanniques a en quelque sorte « accéléré » cette urgence. Désormais, le retrait sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne au 29 mars est, sinon une certitude, tout au moins une véritable possibilité. Le scénario catastrophe du tant redouté, souvent décrit au Royaume-Uni comme un « saut de la falaise », a en effet pris davantage corps avec le vote du Parlement britannique. Or l'échéance du Brexit interviendra, sauf retournement de situation, dans à peine un peu plus de soixante-dix jours, c'est-à-dire demain. Les conséquences d'une sortie sans accord seraient innombrables au niveau tant économique, juridique, financier sécuritaire que géostratégique, ou encore, ne l'oublions pas, Elles restent difficiles à appréhender avec précision, mais il est évident qu'elles seraient absolument considérables, pour Londres en premier lieu, mais aussi pour l'Europe dans son ensemble et la France en particulier, seul pays, je le rappelle, à partager une frontière terrestre, bien que celle-ci soit souterraine, avec le Royaume-Uni. Sans période de transition pour installer la future relation, la rupture serait brutale et aucune mesure de préparation ne permettrait dans ce contexte un Brexit indolore pour l'économie européenne et nationale. Toutefois, il est fondamental que tout ce qui peut être fait pour amortir autant que possible le choc soit entrepris sans délai. L'Union européenne a récemment accéléré ses travaux en la matière et finalise en ce moment même plusieurs mesures de contingence dans ses domaines de compétence. Le niveau national doit naturellement faire de même dans les siens. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera bien évidemment en faveur de ce projet de loi, que l'excellent travail de notre rapporteur Ladislas Poniatowski, très largement repris par les conclusions de la commission mixte paritaire, a par ailleurs permis d'améliorer à plusieurs points de vue. vue. Madame la ministre, permettez-moi de rappeler à cette tribune une évidence : l'adoption aujourd'hui de ce projet de loi n'est en rien un aboutissement, bien au contraire. Je n'ose pas dire qu'il s'agit d'un point de départ, puisque certains pans de la préparation au Brexit ont déjà été lancés ; il s'agit plutôt d'un feu vert du Parlement qui doit permettre au Gouvernement, grâce à ces ordonnances, de déployer tous les moyens et d'entreprendre toutes les actions nécessaires. Je pense bien sûr en premier lieu aux investissements, à la fois humains et matériels, indispensables pour redimensionner et adapter nos systèmes de contrôles douaniers à la nouvelle réalité, notamment dans le domaine sanitaire et phytosanitaire. Il y a encore quelques semaines, notre pays semblait en retard dans ses préparatifs administratifs par rapport à d'autres États comme la Belgique ou les Pays-Bas, ce qui pourrait avoir, pour les régions bordant la Manche et la mer du Nord, des conséquences aussi fâcheuses qu'immédiates en matière de captation de flux commerciaux. Or il est essentiel qu'un éventuel défaut d'adaptation de nos structures, notamment portuaires, n'en vienne pas à constituer un nouveau désavantage compétitif par rapport à nos voisins, qui sont également nos concurrents. À ce titre, le Royaume-Uni a récemment alloué 2 milliards de livres à la préparation d'une sortie sans accord, portant à plus de 4 milliards de livres les fonds destinés aux préparatifs en vue du Brexit depuis 2016. Madame la ministre, pouvez-vous nous livrer une estimation des moyens budgétaires qui seront mobilisés à l'échelon national pour faire face à la nouvelle situation ? Par ailleurs, des efforts considérables devront également être fournis pour mettre en place un accompagnement d'urgence auprès de nos entreprises, qui, pour beaucoup, auront de grandes difficultés à gérer simultanément l'augmentation des droits de douane à venir et l'éventuel changement dans la nature juridique des relations entre l'Europe et le Royaume-Uni. En effet, celles-ci pourraient être bientôt régies mondiale du commerce, l'OMC, et non plus celles du marché unique. Or les récentes déclarations du président du MEDEF International sur l'état de préparation des entreprises françaises sont particulièrement inquiétantes et laissent entrevoir de nombreuses complications. Je le répète, mon groupe soutiendra ce texte qui, malgré les précisions utiles apportées lors de son examen parlementaire, propose toujours des habilitations de portée très générale. C'est pourquoi dans la période tumultueuse qui s'annonce, et pour reprendre la nouvelle rédaction de l'article 4, nous resterons particulièrement attentifs à demeurer informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances, et souhaitons être informés de manière régulière de leur état de préparation. La discussion Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.